La séance est reprise.

Votre gouvernement essaye de minorer la compensation de ce qui constitue la réforme de feue la taxe professionnelle.

On nous parle de la contractualisation pour assainir les finances locales. Nous proposons de revenir sur cette compensation. J'ai lu le rapport de M. Joël Giraud, Giraud, rapporteur général de la commission des finances à l'Assemblée nationale, qui parle de mon département. Samedi, j'ai fait un petit voyage à Neuilly-sur-Seine, monsieur Karoutchi,

Je vous propose d'extraire la dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale et la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, dite DCRTP, des départements de la liste des variables minorées en 2018, sachant qu'elles ont déjà subi une baisse de 12,1 %.

dite DCRTP, des départements de la liste des variables minorées en 2018. Entre la loi de finances initiale pour 2016 et la loi de finances initiale pour 2017, chacun a pu constater une baisse de

des départements de la liste des variables minorées en 2018,

cette diminution de ressources pourrait même être supérieure- c'est le cas de Dunkerque - ou équivalente- comme à Marseille, voire au Havre -à celle de la baisse de la DGF de 2017. Sont tout autant impactées des agglomérations de taille plus modeste et concentrant des difficultés économiques et sociales telles que Denain, Béthune, Maubeuge, Oyonnax,

Après une baisse de 8 % en 2017, soit 34 millions d'euros, ceux-ci seraient ainsi impactés par une baisse de 17 %, soit 66 millions d'euros en 2018. Cette nouvelle ponction des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle aura de nouveau pour effet de pénaliser des communes et groupements de communes défavorisés. Effectivement, ces fonds sont attribués aux collectivités défavorisées selon des critères fixés par chaque conseil départemental, au regard de la faiblesse de leurs ressources fiscales et, ou, de l'importance de leurs charges- je pense notamment à la longueur des voiries, particulièrement dans les territoires ruraux ou de montagne.

par habitant dépassent deux fois la moyenne constatée au niveau national. Le conseil départemental répartit ensuite ces fonds aux communes défavorisées du département selon des critères qu'il fixe librement. Ces fonds permettent à ce titre de renforcer une solidarité nationale envers les communes défavorisées.

La DCRTP est une dotation visant à respecter l'engagement du législateur de garantir qu'aucune collectivité ne soit conduite à voir ses ressources diminuer du fait de la réforme de la taxe professionnelle. Elle est perçue de façon très hétérogène entre les collectivités, et seules celles qui ne bénéficient pas d'un retour CVAE à hauteur de l'ancienne taxe professionnelle en sont Mettre à contribution cette dotation revient donc à pénaliser largement des collectivités déjà fragilisées, alors que les collectivités bénéficiaires nettes de la réforme de la taxe professionnelle ne contribuent pas à cet effort et ne voient aucunement leurs ressources impactées. C'est inéquitable et contre-péréquateur. C'est pourquoi cet amendement vise à supprimer l'élargissement de l'assiette des variables d'ajustement à la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle.

En 2017, le Gouvernement a introduit la DCRTP au sein des variables dites d'ajustement pour financer des mesures de péréquation verticale ou d'exonérations fiscales. La réduction de la DCRTP des régions a été de 8,4 % pour une perte de recettes de 56,4 millions d'euros. L'introduction de la DCRTP au sein des variables d'ajustement est une mesure injuste, inégalitaire, et donc inacceptable pour les régions. cette dotation finance des mesures de péréquation et d'exonérations fiscales qui ne concernent pas les régions. En outre, elle frappe les collectivités pénalisées par la réforme de la taxe professionnelle et qui la perçoivent donc en lieu et place d'une ressource dynamique. Pour 2018, le Gouvernement propose d'appliquer une nouvelle baisse de 6,3 %, ce qui amputerait les recettes des régions de 38,8 millions d'euros. En conséquence, afin d'éviter que les recettes des régions ne soient de nouveau amputées,

Tous ces amendements, cela a été rappelé par M. le rapporteur général, dont je partage nombre des propos sur les difficultés d'estimation du coût et sur les conséquences sur l'équilibre budgétaire,

Si nous intégrons la DCRTP comme nous l'avons fait, cette intégration risque d'amener des collectivités, qui peuvent être fragiles et ont connu la désindustrialisation, à participer au financement de mesures péréquatrices par le jeu des variables de minoration. Je risque de vous décevoir, monsieur le rapporteur général, je n'ai pas aujourd'hui d'amendement à vous proposer, et ce pour une raison bien particulière : le Gouvernement a demandé aux différents services, aux différentes administrations de travailler à la résolution de cette question,

dynamique économique ou industrielle et qui ont retrouvé des activités fortes depuis la réforme de la taxe professionnelle, l'attribution de cette dotation de compensation peut paraître moins justifiée, la fiscalité nouvelle depuis 2010 peut-être plus favorable. Le Gouvernement travaille sur différentes hypothèses, notamment tenir compte du niveau des recettes réelles de fonctionnement, de manière que l'on puisse préserver les collectivités ayant véritablement besoin d'une compensation de la perte liée à la réforme de la taxe professionnelle. Sur la question des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, l'effort qui est demandé cette année est, en termes de progression, non pas inexistant, mais moins important que les années précédentes. L'objectif du Gouvernement est de faire en sorte que

ce jeu permanent du recours aux variables d'ajustement trouve ses limites aujourd'hui. Cela doit nous inciter les uns et les autres à transformer le modèle et le mode de financement des collectivités territoriales. L'avis du Gouvernement est donc défavorable sur l'intégralité des amendements, à l'exception de l'amendement n° I-400, qui permettra de mesurer de manière extrêmement précise, par le rapport qui est proposé, l'impact des décisions prises en matière de fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle.

Le présent amendement vise à majorer la dotation globale de fonctionnement de 180 millions d'euros afin de financer une progression de la dotation de solidarité urbaine, la DSU, et de la dotation de solidarité rurale, la DSR, à hauteur de 180 millions d'euros chacune,

on peut relever une contradiction dans les discours et les comportements. Toutefois, comme disent les philosophes, « la contradiction de la contradiction n'est pas une annulation, mais une locomotive fondamentale de la dynamique. M. Macron, président philosophe, après la philosophie marxiste, vient d'inventer la philosophie « marchiste

les territoires ruraux de développement prioritaires ou dans les zones de revitalisation rurale. Si la connaissance que j'ai de la carte des risques de désertification médicale est encore actuelle, les ZRR et les zones considérées comme des territoires ruraux de développement prioritaires couvrent largement les zones susceptibles d'être classées au nombre des territoires à surveiller. Le dispositif actuel nous paraît

Dans les départements qui anticipent, les difficultés sont très nombreuses, cet amendement va donc dans le bon sens. Au pire, il fera double emploi avec ce qui existe déjà.

et moi-même. Dans notre rapport spécial sur le projet de loi de finances pour 2018, nous avons relevé que les crédits de la dotation d'action parlementaire, dite « réserve parlementaire », destinés aux collectivités territoriales en 2017 n'ont pas été entièrement redéployés. Ces crédits s'élevaient à 86 millions d'euros en 2017, dont 45 millions d'euros provenant de la dotation des sénateurs et 41

le Gouvernement en raison de ses modalités d'attribution. En revanche, son utilité pour soutenir les territoires n'a pas été contestée. C'est pourquoi le présent amendement tend seulement à rétablir les 36 millions d'euros manquants

précise que l'Assemblée nationale a voté un amendement permettant d'affecter 25 millions d'euros à la vie associative, non pas en compensation de la réserve parlementaire, dont vous avez rappelé à juste titre qu'elle avait été supprimée par la loi organique, mais pour continuer à aider les associations. Nous avions également adopté un autre amendement afin

Cette dotation de compensation n'a strictement rien à voir ni avec le problème de l'enveloppe normée ni avec les dotations de l'État et pénalise les communes qui construisent du logement social, alors même qu'on leur demande de le faire.

Nous avons appris que le tribunal d'instance devait transférer 6 347 dossiers, c'est-à-dire l'ensemble des PACS en attente de traitement et des PACS conclus depuis moins de cinq ans, pour lesquels les archives doivent être conservées. En réalité, 7 560 dossiers ont été transférés, car, faute de moyens humains, le tribunal n'était pas en mesure d'extraire les dossiers de PACS dissous depuis plus de cinq ans.

cette procédure en permettant de changer de prénom plus facilement et plus rapidement, sans passer par le tribunal ni faire appel à un avocat. Alors que l'on dénombrait quelque 3 000 demandes chaque année, la déjudiciarisation de la procédure peut contribuer à créer un appel d'air.

afin de garantir aux citoyens un service public de proximité de qualité, cet amendement vise à indemniser les communes qui subissent un nouveau transfert de compétences.

à ce que l'on défalque des éventuelles diminutions de dotations les coûts des charges transférées. Ainsi, il y a deux ans, nous avions proposé de minorer

est à M. le secrétaire d'État. Cet amendement vise à octroyer des compensations au département de Mayotte et aux régions au titre de divers transferts et évolutions de compétences. Ces compensations sont constitutionnellement dues. Plus précisément, son adoption permettra de couvrir les charges résultant de l'alignement des bourses des étudiants en formations paramédicales sur les bourses en vigueur dans les formations universitaires et de la revalorisation de l'indemnité de stage des élèves infirmiers à Mayotte. les charges résultant du transfert des services chargés de la gestion des fonds européens et des agents des centres de ressources, de performances et d'expertises sportives. Est également prévue la compensation des charges afférentes à la troisième année universitaire de mise en place du nouveau diplôme de masseur-kinésithérapeute sous le format LMD, la réévaluation des indemnités de stage des étudiants infirmiers, à l'alignement des bourses des formations paramédicales sur celles des formations universitaires et à la formation professionnelle des détenus

... Il ne faudrait pas que les politiques environnementales, en particulier celles menées par les acteurs industriels ou par les collectivités publiques, soient remises en cause par l'absence de concours financiers permettant de mener un certain nombre d'opérations parfois difficiles à équilibrer. Ainsi, on sait bien que ce sont les concours financiers des agences qui permettent,

en se fondant sur le montant des charges estimé pour l'année suivante. On peut condamner la débudgétisation des actions que permet le financement de ces opérateurs par des taxes affectées, mais plafonner ces taxes ne permet en aucun cas d'améliorer la lisibilité. La rebudgétisation a pour seul effet l'appauvrissement de ces opérateurs, pourtant chargés de missions extrêmement importantes et de plus en plus nombreuses. Depuis le vote de la loi de finances pour 2012, sous l'empire d'un autre gouvernement, la procédure n'a pas été remise en question, variant simplement au fil du temps. nous est offert par le secteur du logement, où nous verrons avant peu que les opérations de construction neuve de logements sociaux ou de réhabilitation du patrimoine existant seront financées par la mutualisation des ressources des bailleurs sociaux. Un peu comme si les locataires du parc locatif social payaient une seconde fois une forme d'impôt sur le revenu pour avoir le droit d'habiter dans un cadre préservé ... Le prélèvement de 2018 sur les ressources de la Caisse de garantie du logement locatif social, c'est 85 à 90 euros d'impôt déguisé par famille locataire du parc social ! Je ne parle pas de la taxe sur les logements sociaux, destinée en principe à l'Agence nationale de l'habitat, opérateur essentiel de la rénovation dans le parc des centres-villes anciens et des copropriétés, mais dont la majeure partie tombe dans les caisses du budget général. C'est donc aujourd'hui le logement qui est visé, comme ce fut hier le secteur culturel, avec les ponctions sur le Centre national du cinéma, par exemple. Le tout, c'est que l'argent vienne alimenter le solde global, à défaut de servir aux usages prévus à l'origine. Cet article de rigueur ne traduit selon nous aucune vision, aucune ambition politique,

Je conviens que la fiscalité affectée peut, dans certains cas, poser un certain nombre de difficultés. Seulement, aller jusqu'à supprimer l'article 19, comme le propose Éric Bocquet, priverait le Parlement

? Il est également défavorable, pour les mêmes raisons. Le mécanisme de plafonnement des taxes affectées a été adopté dans la loi de finances pour 2012 et n'a pas été remis en cause depuis lors. Il permet de piloter un certain nombre de dépenses publiques, notamment des dépenses d'opérateurs ou de divers organismes bénéficiaires des taxes affectées.

à compter du 1 janvier 2018, pour accompagner l'augmentation de la production de chaleur renouvelable en France prévue dans la programmation pluriannuelle de l'énergie- plus 50 % entre 2015 et 2023, soit 6 milliards d'euros d'investissements -et dans le plan Climat du Gouvernement du 6 juillet Mis en place en 2009 par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME, dont le siège est à Angers, le Fonds chaleur s'élève aujourd'hui à 210 millions d'euros. Depuis sa création, ce fonds a aidé 3 988 installations, pour 1,7 milliard d'euros d'opérations d'investissement. Il est proposé de financer cette mesure par un relèvement de la trajectoire de la composante carbone.

les mêmes raisons. Ces amendements sont contraires à la logique de rebudgétisation des moyens de l'ADEME, qui répond à la volonté de renforcer l'effectivité du contrôle parlementaire, ainsi que la maîtrise des recettes et des dépenses publiques. Surtout, cette rebudgétisation s'accompagne d'une consolidation du financement de l'ADEME, puisque ce sont 164 millions d'euros de dotations supplémentaires que l'État allouera à l'agence en 2018 par

ce que nous observons au quotidien dans les territoires, c'est la baisse continue des primes pour épuration. Il s'agit d'un véritable problème pour les communes et leurs syndicats, qui ont besoin de renouveler leur réseau et leurs stations de traitement. Ce que nous observons aussi au quotidien, c'est la baisse régulière des subventions accordées en investissement et les

Plusieurs d'entre nous l'ont déjà évoqué : les agences de l'eau font face depuis de nombreuses années à un élargissement de leurs compétences, avec la biodiversité terrestre, les milieux marins, l'adaptation au changement climatique, qui est un sujet majeur aujourd'hui.

des dixièmes programmes d'intervention, ce qui veut dire que beaucoup de décaissements devront être réalisés dans le cadre d'investissements étalés sur plusieurs années ! Nous sommes raisonnables et équilibrés, pour reprendre le terme employé par le rapporteur général. Nous savons que tous les opérateurs doivent contribuer à l'effort de maîtrise de nos finances publiques.

Ou alors, il faut redéfinir ces missions, et c'est au Gouvernement de le faire ! Je propose un amendement raisonnable, qui a d'ailleurs été adopté par la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat.

concernant les agences de l'eau de 2018 à 2019, mais de maintenir en 2018 un prélèvement identique ou quasi identique à ceux qui ont été opérés en 2015, 2016 et 2017. Le rapporteur général vient de déclarer que le maintien de ce prélèvement au titre de l'année 2018 paraissait

pour explication de vote.

que les différentes mesures prises auraient pu ou devraient se traduire par une diminution du coût incombant à l'usager. Dans le même temps, un certain nombre de parlementaires ont indiqué que, dans le cadre

pourtant à accepter la réduction de 20 millions d'euros pour 2019. On ouvre la discussion, on met tous les sujets sur la table et, ensuite, seulement on décide.

De deux choses l'une : ou l'argent du CNDS sert à développer les pratiques sportives de masse et, dans ce cas, l'effort destiné au haut niveau est assumé par le budget général, ou alors, on réduit la quotité des enjeux rétrocédés au Centre pour faire de la Française des jeux une bonne affaire pour quelque acheteur potentiel d'avenir Une telle démarche visant à priver de plusieurs milliers d'euros la pratique sportive de proximité ne nous semble pas la meilleure voie à suivre. Rassurez-nous, monsieur le secrétaire d'État, et préservez l'intégrité des ressources du CNDS !

par le maintien des plafonds actuels pour le prélèvement de 1,8 % sur les paris sportifs, pour le prélèvement exceptionnel de 0,3 % sur les jeux d'argent et de hasard et pour la taxe « Buffet » sur la cession des droits télévisés sur les événements sportifs en France, par le maintien des plafonds actuels pour le prélèvement, ainsi qu'une modification du plafond sur le prélèvement principal de 1,8 % sur les jeux. Les moyens du CNDS économisés- hors rebudgétisation -sont ainsi intégralement maintenus, afin de lui permettre de poursuivre ses missions essentielles au service du sport pour tous, dans la perspective des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

de mauvaises surprises sur des sommes tout de même extrêmement importantes.

quelques précisions pour la bonne compréhension de nos débats. L'article 19 prévoit d'abaisser de 150 millions d'euros le plafond de la taxe affectée aux CCI,

assujetti à la taxe pour frais de chambre consulaire et comme il s'agissait d'une entreprise publique, une disposition de la loi de finances pour 2010 avait prévu que le montant de la taxe acquittée serait directement reversé

les chambres de commerce et d'industrie ont subi depuis quelques années une ponction extrêmement forte, qui les a contraintes à se réorganiser totalement et a placé bon nombre d'entre elles dans une très grande difficulté financière.

les conséquences sur l'investissement dans les territoires, notamment au niveau des centres de formation et d'apprentissage, ainsi que sur le fonctionnement interne des chambres consulaires. Je prendrai l'exemple de la chambre de commerce et d'industrie de Paris Île-de-France, dont la baisse des ressources fiscales représente une perte de 37 millions d'euros. Entre 2015 et 2016, 1 000 collaborateurs agents publics sont partis, soit 20 % des effectifs. La conséquence immédiate, c'est une baisse des investissements dans les écoles gérées par la chambre de commerce et d'industrie, investissements représentant 60 % du budget. Ce sont ainsi 19 établissements d'enseignement et de formation dans 8 départements

nous avons besoin de ces investissements dans les centres d'apprentissage et dans les grandes écoles prestigieuses qui sont financées par les chambres de commerce et d'industrie, notamment celle de Paris Île-de-France. C'est pourquoi, mes chers collègues, je vous propose de voter cet amendement, tendant à supprimer la baisse du plafond pour l'année prochaine. Les

nombreux contacts avec des entreprises, ont pu constater combien il est difficile de faire coïncider l'offre et la demande d'emplois dans notre pays. Les outils consulaires, par leur implication dans le domaine de la formation, permettent justement cette adéquation. Ils offrent une réponse aux besoins des entreprises

La baisse de la ressource fiscale des CCI prévue dans cet article 19 du projet de loi de finances fait courir un risque important aux finances de certaines CCI dans l'Hexagone, mais singulièrement dans les outre-mer. Cette baisse unilatérale de la fiscalité affectée touchera effectivement les CCI dans leur globalité, sans tenir compte de leur situation financière ou de leurs actions. Si l'on ne prend que l'exemple des CCI des outre-mer, mais des exemples similaires peuvent être trouvés ailleurs, le volume financier, entre 2010 et 2015, est passé de 300 à 117 millions d'euros pour les quatre départements après la perte des concessions dont la rémunération alimentait le budget général des CCI. Celles-ci connaissent aujourd'hui d'importantes difficultés financières, que ne traduit pas, certainement, certainement, la simple analyse de leurs taxes affectées. C'était d'ailleurs la raison qui avait poussé le Président de la République à prendre pour engagement de campagne qu'elles ne seraient plus concernées par une éventuelle baisse des ressources. Cet engagement semble remis en cause par cet article 19. Puisque le ministère des finances a pris l'engagement que cette baisse de la fiscalité affectée serait la seule du quinquennat, nous proposons qu'elle soit étalée sur la durée de ce quinquennat, afin de donner aux CCI le temps de trouver une solution plus fine et de les accompagner dans leurs réformes, sans impact à terme sur les finances publiques. La

Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement est un peu différent des précédents, comme l'a indiqué M. le rapporteur général. Une réduction aussi drastique des crédits conduira évidemment à s'interroger sur les fonctions qui doivent être assurées par le réseau consulaire. nos structures publiques d'accompagnement des entreprises sont aujourd'hui au milieu du gué : plusieurs réseaux consulaires, plusieurs opérateurs publics, plusieurs collectivités territoriales assurent chacun une fonction d'accompagnement auprès des entreprises françaises sur notre territoire, comme à l'étranger, sans que leurs actions soient pour autant suffisamment coordonnées et complémentaires pour éviter les redondances. Cette situation est non seulement préjudiciable aux finances publiques, mais surtout aux entreprises elles-mêmes, qui peuvent peiner à trouver l'interlocuteur le plus pertinent et, en tout état de cause, ne bénéficient pas du de prestations à même de les aider efficacement dans leur création, puis leur développement. C'est donc plus largement tout l'écosystème de l'accompagnement public des entreprises qu'il faut questionner et, probablement, repenser. Or cette réflexion, pour être fructueuse, nécessite du temps et l'on ne saurait s'y engager de manière raisonnable en mettant à mal l'exercice immédiat des compétences de l'un des réseaux.

qui consiste à augmenter la part faisant l'objet d'une péréquation dans les recettes affectées aux chambres de commerce et d'industrie. En un mot, il a été rappelé que la trésorerie globale des CCI s'élevait à environ 500 millions d'euros. Lorsque l'on compare les 150 millions d'euros de prélèvement à ces 500 millions d'euros de trésorerie, les chiffres peuvent sembler sans commune mesure, sauf que cette trésorerie globale cache des disparités

est donc bien évident que, sans un minimum de trésorerie, elles ne pourraient plus fonctionner. Or, comme je l'ai dit tout à l'heure, elles sont absolument indispensables pour permettre le développement des dispositifs de formation professionnelle,

me rallier au panache du rapporteur général

de métiers et de l'artisanat. En l'occurrence, c'est particulièrement injuste parce que ces dernières ont fait de gros efforts pour rationaliser leur action.

du geste professionnel- c'est absolument essentiel - ; faire du numérique un outil incontournable de l'adaptation de l'entreprise artisanale. Malgré cela, elles sont quand même ponctionnées. J'aimerais rappeler les sages paroles du président Macron Je souhaite mettre dès le début du quinquennat une stratégie claire en place : je vais mettre fin à la régulation annuelle budgétaire qui conduit au rabot.

Cet amendement a pour objectif de sauvegarder les dispositions de l'article 41 de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

monsieur le rapporteur

des chambres de métiers et de l'artisanat devrait s'élever à 39,89 millions d'euros, alors que la collecte s'élèverait, hors contribution des micro-entrepreneurs, à 43,5 millions euros, soit un écrêtement de près de 3,6 millions d'euros.

relatifs à des dispositions visant à rétablir le plafonnement des contributions des chefs d'entreprise immatriculée au répertoire des métiers au titre de la formation professionnelle, à la fois perçues par le FAFCEA et par les chambres de métiers et de l'artisanat, au titre des conseils de la formation qui n'interviennent que sur les formations en gestion et transversales. Cet amendement a pour but de sauvegarder les dispositions de l'article 41 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. article permet de déplafonner, à compter de 2018, la contribution à la formation professionnelle des chefs d'entreprise immatriculée au répertoire des métiers, versée au FAFCEA et aux chambres de métiers et de l'artisanat au titre des conseils de la formation. Ce déplafonnement est motivé par le fait que la contribution à la formation professionnelle finançant des droits sociaux individuels ne doit pas être limitée pour une seule partie des travailleurs indépendants, en l'occurrence les artisans. de l'article 41 est de sanctuariser l'intégralité de l'effort contributif des artisans à leur formation et d'assurer la pérennité de la ressource qui finance leurs droits, en cohérence avec l'extension du compte personnel de formation.

71 millions d'euros en 2018 -afin de faire mettre en oeuvre par l'État un renforcement des actions de prévention, en particulier pour les risques d'inondation et de submersion marines. À l'heure de la concertation pour la création d'un second plan d'adaptation au changement climatique qui mettra l'accent sur l'importance de la prévention face aux risques dévastateurs liés à celui-ci, il paraît incompréhensible que la France fasse le choix d'affaiblir financièrement un secteur aussi stratégique pour l'avenir. Comment, à l'heure où la prévision et la prévention peuvent être les rares armes dont nous disposons pour éviter des catastrophes humanitaires à la chaîne, la France peut-elle manquer d'ambition au point de se démunir d'une capacité d'investissement sur l'avenir ? Mes chers collègues, tous les territoires sont aujourd'hui attentifs à leurs capacités de résilience face aux aléas climatiques, dans tous les domaines- inondations, incendies, sécheresses, etc. Amputer le Fonds de prévention des risques naturels majeurs serait un signal décourageant face à la nécessité d'une mobilisation totale et continue des collectivités sur ce sujet. L'État doit

du rapporteur spécial- ici présent -sur le compte de concours financiers « Avances à l'audiovisuel public », qui a considéré que la diminution des ressources de France Télévisions constitue un premier pas nécessaire dans l'attente d'une réforme d'ensemble du secteur audiovisuel public. Cette réforme est annoncée par le Gouvernement pour 2018, et vous savez que les années

ou assurer une solidarité financière avec les chambres territoriales de leur ressort en difficulté. Le texte adopté par l'Assemblée nationale prévoit de presque doubler son montant, en le fixant à un maximum de 40,5 millions d'euros. Ce mécanisme de péréquation financière ne doit pas se retourner contre les chambres qui, depuis plusieurs années, ont entamé des actions de restructuration de leur réseau et réduit leurs dépenses corrélativement à la forte baisse des financements publics depuis 2012. Il serait en effet plus que souhaitable que ce fonds de péréquation puisse accompagner ces chambres qui, à nouveau, compte tenu de la baisse du plafond de la taxe affectée prévue pour 2018, devront aller encore plus loin dans leur réorganisation et dans la suppression de certaines de leurs activités en faveur des entreprises ou dans le domaine de la formation et de l'enseignement. lors, cet amendement vise à flécher un tiers des sommes mobilisées dans le cadre du fonds au profit des CCIR qui ont réalisé des efforts de rationalisation et de mutualisation substantiels.

d'industrie prévoient des dispositifs de péréquation et de solidarité financière. En particulier, un montant est versé aux CCIR pour financer des projets structurants de modernisation des chambres ou contribuer à la solidarité financière. Les dispositions et les débats à l'Assemblée nationale ont permis d'augmenter la part consacrée à la péréquation. Le fonds de péréquation mis en

Par ailleurs, ces projets sont autant de projets de mutualisation et de rationalisation qui visent notamment à améliorer l'offre des chambres de commerce et d'industrie tout en diminuant les coûts. Il serait donc paradoxal d'accorder, dans la possibilité de financer ainsi ces projets, une forme de priorité à ceux qui ont déjà pu mener de tels projets de réduction des coûts. Enfin, j'ajoute que la définition

pour vérifier que les économies envisagées ont été réelles, ensuite parce que de nombreuses chambres régionales ont été créées au 1 janvier 2017, notamment dans les Hauts-de-France, en Auvergne-Rhône-Alpes, dans le Grand Est, en Nouvelle Aquitaine, et que le calcul de la diminution des coûts afférents n'est pas aisé à réaliser à ce stade. Madame Lamure, l'amendement n° I-95 est-il maintenu

un critère d'accès à la part de péréquation, qui est celui de la part des communes classées en ZRR dans le ressort de la chambre de commerce et d'industrie, par un critère de densité démographique. Dans la mesure où le classement du territoire en ZRR tient compte d'un certain nombre d'éléments, notamment l'activité économique, le niveau de revenu des habitants et le niveau d'activité des entreprises, il nous paraît plus opportun de maintenir le critère ZRR

qui est non seulement inutile, mais introduit du risque et de la complexité. L'alinéa 46 de l'article 19 conditionne le bénéfice du fonds de péréquation pour les chambres de commerce et d'industrie infradépartementales dont le périmètre comprend au moins 60 % de communes ou de groupements de communes classés en zone de revitalisation rurale à la mise en oeuvre d'un processus de fusion avant le 1 août de chaque année.

L'effort de rationalisation qui se cache derrière cette nouvelle disposition est déjà engagé. Nous savons bien que les réseaux consulaires ont d'ores et déjà mis en oeuvre de nombreux efforts pour engager des mutualisations territoriales ont déjà été supprimées en trois ans. Parallèlement, le classement en ZRR est évolutif. Forcer des chambres de commerce et d'industrie infradépartementales dont le périmètre comprend au moins 60 % de communes classées en ZRR à fusionner, c'est oublier que que le classement ZRR évolue et se réforme, nous le savons bien, chers collègues. C'est donc introduire un risque, une complexité, une suspicion pour des territoires et des bassins économiques qui portent des projets de long terme et ont un besoin de visibilité pour construire. L'article 1600 du code général des impôts que l'article 19 propose de modifier est suffisamment complexe. Les chambres de commerce et que les règles encadrant le fonds de modernisation et de péréquation des chambres de commerce et d'industrie soient maintenues en l'état du droit actuel et que les montants et règles d'affectation du fonds de modernisation et de péréquation ne soient pas modifiés. Un fragile équilibre a été obtenu sur le fonds de péréquation et de modernisation au cours des deux dernières années. Je crois donc, mes chers collègues, qu'il faut faire confiance aux acteurs économiques du territoire qui sont à même d'apprécier les périmètres des bassins d'emplois. Il ne faut plus les pénaliser,

du Gouvernement ? Cet amendement vise à supprimer la condition d'éligibilité introduite par un amendement du rapporteur général de l'Assemblée nationale au bénéfice du fonds de péréquation pour les chambres de commerce et d'industrie qui sont engagées dans un processus de fusion.

ses propres modalités de financement. L'une des pistes évoquées est la mise en place d'une contribution volontaire obligatoire de manière à ce que les acteurs du commerce et de l'artisanat puissent, sans avoir recours à une taxe affectée, élément de fiscalité publique,

parole est à Mme Annie Guillemot. Le Fonds national des aides à la pierre, le FNAP, a été créé en 2016. Il est chargé de gérer les aides à la pierre et d'associer plus étroitement les collectivités locales à la production de logements sociaux. Le principe retenu était celui d'un d'un financement paritaire entre État et bailleurs sociaux. Or le projet de loi de finances pour 2018 prévoit d'augmenter la contribution des bailleurs sociaux de plus de 100 millions d'euros, en la portant de 270 à 375 millions d'euros. Dans le même temps, pour 2018, la contribution de l'État tombe à 50 millions d'euros au lieu de 200 millions d'euros en 2017, soit 150 millions d'euros millions d'euros de moins. Le désengagement de l'État des aides à la pierre est un très mauvais signal : il rompt le pacte fondateur conclu entre l'État et les bailleurs sociaux, fondé sur le principe du financement paritaire du FNAP par l'État et les bailleurs sociaux. Cette mesure, ajoutée à la décision du Gouvernement de baisser de 1,5 milliard d'euros les APL dans le parc public, va totalement remettre en cause le modèle social et républicain du logement social en France. Il s'agit donc de maintenir, pour 2018, la contribution des bailleurs sociaux au FNAP au même montant que celui de 2016 et 2017, soit 270 millions d'euros. Quel est l'avis de la commission ? Je ne veux

de nombreuses formes de coopération existent entre les collectivités territoriales et les chambres consulaires afin d'assurer un développement pragmatique des territoires, un soutien aux filières innovantes et la promotion des savoir-faire, le le projet de réduction du nombre de chambres de commerce ou des chambres de métiers risque d'entraîner une dégradation du service de proximité de soutien aux entreprises. La rédaction d'un rapport ne répondant pas à la problématique posée, il semble préférable de supprimer l'alinéa 65 ajouté par l'Assemblée nationale.

Cet amendement tend donc à recentrer ce rapport sur les évolutions possibles au sein de chacun des deux réseaux et sur les pistes de coopération qui pourraient être développées au service des entreprises et des territoires. L'artisanat est un secteur économique dont les spécificités exigent le maintien d'un réseau consulaire dédié à l'accompagnement de ses entreprises et à la formation aux métiers par l'apprentissage. Les neuf amendements suivants

de nombreux territoires. J'ai assisté ce matin, je l'ai dit tout à l'heure, à l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat du Finistère. Il a été rappelé que toutes les institutions consulaires fonctionnent ensemble. Une conférence économique des chambres consulaires existe dans le département. Là où c'est possible, les locaux sont mutualisés entre les différentes institutions consulaires. D'autres projets sont en préparation, mais ils ne doivent pas conduire

consulaire et sur les pistes de coopération qui pourraient être développées entre les deux réseaux, au service des entreprises et, surtout, des territoires.

J'avais déjà présenté cet amendement l'année dernière. Nous en revenons aux taxes affectées. Je vous propose de diminuer les tarifs de la taxe de solidarité sur les billets d'avion de sorte que son produit

Cet amendement vise à améliorer l'information du Parlement sur le volume et la dynamique de la fiscalité affectée à des opérateurs, cinq ans après le rapport du Conseil des prélèvements obligatoires. Ce rapport avait permis un premier aperçu de l'ampleur de ce phénomène, qui contrevient au principe de l'universalité budgétaire. Une revue quinquennale pourrait permettre de faire le point sur les mesures déjà adoptées et sur l'opportunité de renforcer l'encadrement des taxes affectées. Quel

du stock très important de navires- on parle de 35 000 - en attente de déconstruction. Le Gouvernement sera au rendez-vous pour y affecter les crédits nécessaires,

Sur 250 000 navires taxables, y compris ceux dont le montant du droit est au-dessus ou au-dessous du seuil de perception et les navires exonérés, seulement 90 000 sont effectivement taxés taxés en 2017. Selon les chiffres recensés en 2016, les 10 000 navires de moins de dix ans contribuent à hauteur de 16,5 millions d'euros au produit brut du DAFN, tandis que les 160 000 navires de plus de vingt-cinq ans n'y contribuent qu'à hauteur de 5 millions d'euros. Il serait souhaitable d'en

Actuellement, le code forestier ne considère pas les opérations portant sur les plantations de chênes truffiers comme un défrichement. Ces opérations sont ainsi dispensées d'autorisation préalable et sont également dispensées des obligations auxquelles sont soumis les défrichements, comme des replantations ou le paiement d'une indemnité de compensation. Paradoxalement, si un trufficulteur souhaite défricher un bois pour planter des chênes truffiers, il est soumis aux obligations énoncées ci-dessus, notamment le versement d'une indemnité compensatoire, destinée à alimenter le Fonds stratégique de la forêt et du bois et dont le montant représente environ 3 000 euros par hectare. Le paiement de cette indemnité, outre son incohérence, constitue un frein majeur au développement de la trufficulture dans les territoires ruraux et peut avoir pour conséquence l'annulation de projets de plantation. Il est donc indispensable de la supprimer. Il est également important de signaler que cette indemnité perdure dans un contexte où la France importe près de 80 % des truffes consommées en France- nous en produisons seulement 20 %. Par ailleurs, cette production constitue dans bien des cas une activité complémentaire pour les agriculteurs et s'inscrit dans une démarche intéressante de diversification. Enfin, le développement de truffières concourt à la préservation de la biodiversité, car elles jouent un rôle de refuge pour de nombreuses espèces d'êtres vivants.

La loi de finances pour 2018 prévoit à l'article 19 une nouvelle baisse très importante des ressources affectées aux CCI, d'un montant de 150 millions d'euros. Afin de préserver l'outil des CCI et sa performance sur tout le territoire, il apparaît indispensable de trouver des sources financières de compensation. Or le 5.3.5 de l'article pour 2010 a institué un prélèvement au profit de l'État sur les ressources de la TACFE affectée à l'origine par France Télécom-Orange aux chambres de commerce et d'industrie. Ce prélèvement a été maintenu depuis, sans fondement. Il s'élève chaque année à 28,9 millions d'euros. Cet amendement propose de supprimer une telle disposition, qui constitue un prélèvement masqué sur les entreprises, contribuant à accroître les ressources de l'État et non à financer les actions menées par les CCI au service de ces mêmes entreprises. Il convient de noter que supprimer ce prélèvement rendrait ainsi 28,9 millions d'euros aux CCI sans accroître la fiscalité sur les entreprises, puisque cette somme est bien versée par France Télécom-Orange, et sans toucher au plafonnement de la TACFE. L'amendement permet ainsi de compenser légèrement la baisse de ressources fiscales prévue par le Gouvernement.

l'amendement n° I-197. Cet amendement vise à supprimer une anomalie, à savoir le prélèvement dit France Télécom sur les ressources fiscales des CCI. Ce prélèvement visait à rembourser l'État de la taxe pour frais de CCI qu'il déboursait pour France Télécom, l'État considérant que, compte tenu du fait qu'il en était actionnaire référent, France Télécom n'aurait pas dû avoir à s'acquitter de cette taxe. Néanmoins, depuis la privatisation de France Télécom en 2004, ce prélèvement n'a jamais été supprimé, il a même été pérennisé, en étant reconduit dans la loi de finances pour 2010. Il s'agit pour l'État d'un mode de prélèvement sur les entreprises invisible pour le grand public, puisqu'il se fait au détriment des CCI. À l'heure où nous demandons d'importants efforts financiers au réseau des CCI et où nous les incitons à se moderniser et à se rationaliser, il me semble que l'État doit aussi mettre fin à ce type d'anomalie, en supprimant ce prélèvement. Tel est l'objet de cet amendement.

Chaque année, France Télécom-Orange s'acquitte, comme toutes les entreprises, de sa taxe pour frais de chambre. Toutefois, la somme versée ne fait que transiter dans les comptes des CCI, puisqu'elle est reversée automatiquement au budget général de l'État pour un montant annuel de 28,9 millions d'euros. Ce dispositif est appelé « prélèvement France Télécom ». Il se justifiait, en son temps, par le fait que France Télécom était une entreprise publique. Il n'a aujourd'hui plus aucun fondement juridique et constitue simplement une ponction supplémentaire de l'État sur les ressources affectées

Pour compenser en partie cette baisse et préserver les capacités d'action des CCI, une source de financement existe, puisqu'une partie des ressources de la TACFE est aujourd'hui affectée à l'État, alors qu'elle était à l'origine versée par France Télécom aux CCI. Cette affectation s'élève à 28,9 millions d'euros par an. Cet amendement propose de revenir à la situation qui prévalait avant la loi de finances pour 2010, en allouant à nouveau ce prélèvement directement aux CCI.

est ainsi libellé : La parole est à M. Olivier Cadic. L'article 137 de la loi de finances pour 2016, modifiant l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003, a créé une taxe pour le développement des industries de la transformation des matières plastiques. Lorsque des entreprises d'un même groupe se vendent des produits soumis à la taxe, celle-ci s'applique à chaque vente. Dans le secteur de la plasturgie, une filiale peut vendre un semi-produit à une autre filiale ou à sa société mère qui, à son tour, le transformera, peut-être, avant de faire de même, jusqu'au produit final mis sur le marché. En conséquence, le produit final, qui a pu faire l'objet de plusieurs transferts au sein d'un même groupe, est donc taxé plusieurs fois, ce qui crée une distorsion de concurrence pénalisant sans raison certaines entreprises au seul motif de leur organisation juridique interne. De plus, les importations en provenance de l'Union européenne étant exonérées de la taxe, il est plus intéressant, dans un groupe, d'acheter les semi-produits à des filiales situées au sein de l'Union européenne, hors France, qu'en France où la vente est taxée. Cette situation porte préjudice sans raison aux entreprises françaises face à leurs homologues situés dans le reste de l'Union européenne. L'objet de cet amendement est de corriger cet effet de bord non souhaité en rendant impossible l'application en cascade de la taxe,

L'Union européenne a fixé un objectif de 95 grammes d'émissions de dioxyde de carbone par kilomètre pour les véhicules à l'horizon de 2020. Cet objectif a été repris par le Gouvernement : le ministre de la transition écologique et solidaire l'a inscrit dans son plan Climat, et le chef de l'État a rappelé cet engagement tout récemment à Berlin.

le moins toxique pour la santé, et encore moins à aller vers des motorisations propres. En différenciant les deux sources de carburant et en établissant une certaine équité entre l'essence

n'a pas pu valider l'abaissement à 115 grammes, en faisant référence à la cohérence avec un autre texte. Or cet autre texte, c'est celui qui est en débat aujourd'hui. C'est donc le moment, monsieur le secrétaire d'État, non seulement de faire acte de cohérence avec les engagements pris, mais aussi de rendre service à votre collègue ministre de la santé en actant la diminution à 115 grammes des émissions de CO2 dans le calcul du malus automobile. Quel est l'avis de la commission ?

un alourdissement de la fiscalité sans augmentation des recettes dont bénéficie France Télévisions, puisque celles-ci seraient limitées par le plafonnement. En cohérence avec ce que j'ai dit tout à l'heure et en attendant la réforme globale, j'émets un avis défavorable. M. David Assouline, pour explication de vote.

Restons cohérents ! Le service public de l'audiovisuel a largement de quoi fonctionner en 2018. Attendons les propositions de réorganisation et, à ce moment-là, nous aurons un débat serein sur le financement, en fonction de la réorganisation

Nous faisons avec M. Vaugrenard une autre proposition, qui a déjà été présentée dans cet hémicycle et qui m'apparaît parfaitement réaliste. Tout le monde sait qu'il faut augmenter les ressources de France Télévisions.

mais cette extension aux résidences secondaires au sein desquelles il y a une télévision apporterait la ressource que nous recherchons. Je sais bien qu'elle

La taxe d'habitation va être supprimée, en tout cas pour certains contribuables, par dégrèvement et en trois ans, avec l'objectif de 80 % de contribuables exonérés. Nous sommes, je crois, à peu près tous convaincus qu'un impôt qui ne serait payé que par 20 % des contribuables n'est plus un impôt acceptable. Le véritable horizon de cette réforme, que je souhaite, est une réforme fondamentale de la fiscalité locale. Le Président de la République a invité

un pool de reporters à l'étranger qui nous permettent de faire encore exister une information puisée par le service public à l'étranger. Le tout dans un environnement concurrentiel qui va nous détruire. À l'inverse d'autres services publics,

d'une disposition de cet article, aux termes duquel l'État va emprunter 1,7 milliard d'euros pour les prêter au consortium privé qui doit réaliser le Charles-de-Gaulle Express.

Dans le même temps, l'État est en train de nous expliquer que la société du Grand Paris ne va pas pouvoir réaliser la ligne 17 du métro automatique, qui doit aussi aller jusqu'à Roissy-Charles-de-Gaulle, et même au-delà, jusqu'au Mesnil-Amelot,

est en cause, ce n'est pas le financement de la ligne, puisque le modèle de financement de la SGP est robuste : 500 millions d'euros de ressources lui sont affectés chaque année. On peut donc parfaitement réaliser cette partie de la ligne de la SGP

qu'on refuse de réaliser la ligne 17 du métro automatique, porteuse d'avenir, porteuse d'investissements et de richesses pour le pays. Je l'admets d'autant moins que, dans le même temps, l'État va prêter 1,7 milliard d'euros au consortium qui va faire le Charles-de-Gaulle

par une forme de déficit public. En effet, le budget de l'État n'étant pas en excédent, ce prêt sera forcément de nature à aggraver le déficit public au sens maastrichtien du terme. Pourquoi le Gouvernement a-t-il choisi

considérés même comme instables et qui ne semblaient pas assez solides pour pouvoir être totalement mis en oeuvre. C'est la raison pour laquelle, de manière très exceptionnelle- M. le rapporteur général a raison -, l'État a préféré passer par

est juste. Il connaît son territoire et la difficulté grandissante et journalière de tous ses concitoyens et concitoyennes à utiliser les transports dans cette partie de l'Île-de-France.

que fait le Gouvernement, c'est finalement d'aller dans le sens d'Aéroports de Paris, qui veut dissocier les passagers quotidiens que nous sommes

de toutes ces personnes qui prennent les transports dans des conditions insupportables et inhumaines. Merci pour votre amendement, monsieur

la ligne Charles-de-Gaulle Express et l'état du réseau. Il faut trouver plus de moyens pour le réseau, et la région, aujourd'hui, s'y consacre beaucoup. Je regrette qu'on ait

pour aller jusqu'à Roissy, ils auront payé pour rien ! Le deuxième projet qui nous importe, c'est l'interconnexion avec la ligne H- la principale ligne du Francilien, qui dessert le Val-d'Oise radialement vers Paris.

une réponse intéressante sur la réalisation de l'ensemble du métro prévu au titre du Grand Paris. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

se terminer. À force de mettre sur la table tellement de projets de transport qui coûtent si cher, l'État va être obligé de faire des choix. Or comment vont être dictés ces choix ?

donc : ne remettons pas en cause le Grand Paris Express ! Finançons le Charles-de-Gaulle Express si nous en avons la capacité, mais ne faisons pas l'un au détriment de l'autre